La séance est ouverte, le compte rendu analytique de la présente de la précédente séance a été distribué, il n'y a pas d'observation, le procès verbal est adoptée sous les réserves d'usage. La parole est à madame Valérie Létard, pour une mise au point sur un vote. Merci monsieur le président, chers collègues, lors du scrutin public numéro 44 du 13 décembre 2017 portant sur l'ensemble de la proposition de résolution en application de l'article 34 de la Constitution relatives au développement du fret ferroviaire, monsieur Bernard Delcros a été compté parmi les personnes votant contre, il souhaiterait rectifier son vote et voter pour cette raison, cette résolution, je vous remercie. Merci, cher collègue, donner de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution visant à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission, présenté par Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Philippe Bas, rapporteur de la commission des lois, et néanmoins président de ladite commission. Monsieur le président, merci de me donner la parole monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs sert collègues je suis heureux de vous présenter cette résolution préparée par Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat et qui vise tout simplement à conforter une expérimentation que le Sénat avait lancé dont il avait pris l'initiative d'expérimentation de la législation en commission le terme peut paraître exagéré, car c'est bien sûr l'assemblée elle-même qui adopte le texte de loi qui font l'objet de cette procédure. Le Sénat, à cet égard, a su innover et si au mois de juillet dernier, le président de la République a souhaité que cette procédure puissent être mises en oeuvre dans les 2 assemblées, nous n'avons plus que nous réjouir de Ferraci école en n'aspirant des réformes plus larges sur ce point, la procédure de législation en commission à jouer à 6 reprises pour 4 textes, dont 2 textes de loi organique, elle permet de délibérer en commission mais publiquement et en présence d'un membre du gouvernement d'un certain nombre de textes chacun. De nos collègues non membres de la commission peut participer aux travaux de la commission dans le cadre de cette procédure, mais seuls les membres de la commission, vote sur les amendements qui sont soumis à leur appréciation le texte élaboré par la Commission vient ensuite en séance, il donne lieu à une discussion générale et sauf exception circonscrite par notre règlement, il ne donne pas lieu amendement en séance pour apporter la garantie que cette procédure ne se généralise pas car la règle commune, ça doit rester évidemment le débat dans l'hémicycle et la discussion des amendements dans l'hémicycle un droit de véto est prêt. La procédure de législation en commission est en effet décidée par la conférence des présidents

pour éviter la généralisation de ce type de procédure qui est extrêmement utile dans certains cas et qui pourrait, dans le cas de textes très importants, être au contraire préjudiciable au bon fonctionnement du parlement et à la libre expression de chacune et de chacun d'entre vous pour la défense de ses amendements dans l'hémicycle, lui-même ce droit de véto ne peut peut être exercée, non seulement au moment où la conférence des présidents se prononce sur l'application à texte donné de la procédure de législation commission mais il peut aussi être utilisée par le président du groupe. La réunion de la commission comme laquelle le texte de la Commission a été adopté, autrement dit on peut démarrer la procédure avec l'application du système de législation en et l'arrêter en cours de route pour reprendre le cours normal du débat sur le texte de loi soumis à l'examen de notre assemblée, c'est bien qu'on peut imaginer d'ailleurs que si telle ou telle mécontents du texte de la commission, il aura une seconde chance après la réunion de la commission pour que tout soit remis en jeu devant notre assemblée, je crois que c'est garanti sentent très importante, on pourrait, et ça a été le cas au cours de certaines des auditions que j'ai tenus pour préparer mon rapport, certains voudraient qu'on aille plus loin, mais il n'y aurait pas de consensus entre nous pour le faire et sur un sujet qui concerne chacune et chacun d'entre nous, il est bon tout de même que, même si ce projet de résolution ne sera probablement pas votée par les membres de tous les groupes, il y a au moins un consensus minimum, je crois que les concertations auxquelles le président du Sénat, a procédé, les auditions qui ont suivi, permettent de garantir ce minimum de consensus sur lequel la réforme ne serait certainement pas souhaitable, qu'il y a eu une novation par rapport au système que nous avons expérimenté pendant 3 ans, c'est que, désormais, si vous adopter cette résolution qui modifie notre règlement, nous pourrons scinder un texte en plusieurs parties, une partie qui sera examiné selon la méthode de la législation en commission et une autre partie, il faudrait bien sûr que, elle puisse être totalement distinguer du reste du texte, qui serait discutée selon la voie normale, nous verrons si nous inscrivons cela dans notre règlement, dans quelle mesure cela correspondra réellement un besoin en tout cas la faculté nous serait ouverte, ce qui m'a paru être plutôt une bonne chose, voilà, mes chers collègues, la présentation que je voulais faire de cette réforme, qui montre que le Sénat continue à aller de l'avant, quand il s'agit de moderniser ses méthodes de travail. Merci beaucoup, une président. à la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Yvon Collin. Pour le groupe RDSE et pour 6 minutes chers collègues. Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des lois sur le rapporteur, chers collègues, en d'autres circonstances, l'annonce d'une proposition de modification de notre aveuglement précédent une réforme constitutionnelle rit plus paraître incongrue, la logique voudrait que l'on adapte le règlement d'eau modifications introduites par les lois constitutionnelles ou des lois organiques, plutôt que l'inverse, pourtant dans le contexte continue d'un affaiblissement institutionnel du Parlement face à l'exécutif et à l'approche de la prochaine révision constitutionnelle, cette démarche est la bonne, les députés emboîter également le pas après la publication hier du compte rendu des groupes de travail sur la réforme du fonctionnement de l'Assemblée nationale, leur proposition numéro 6 intitulé simplifier l'examen des textes les plus consensuelles, en prévoyant un examen uniquement commission reconnaît d'ailleurs explicitement l'avancée de la réflexion sénatorial en la matière ces hommages sens suffisamment rare de la part de cette assemblée pour être souligné, c'est pourquoi nous soutenons la proposition de résolution du président Larché, elle illustre d'ailleurs la capacité d'initiative de notre haute assemblée et notre volonté de prendre une part active à l'élaboration de la future réforme constitutionnelle après la dernière modification de la Constitution n'est plus de 25 ans après la publication d'un rapport du Conseil d'État condamnant entre guillemets les bavardages de la loi, les critiques contre le Parlement n'ont guère évolué, le renforcement des commissions permanentes dans la procédure législative, à l'évidence n'a pas permis d'en faire disparaître les causes, comme nous l'avions anticipé à l'époque, à l'inversion de la règle selon laquelle le texte examiné en séance publique, est désormais le texte adopté en commission et non plus le texte initial face aux successives, tentative de rationalisation de la procédure législative, notre position est toujours restée constante, celle de rappeler le rôle déterminant du Parlement en faveur des libertés et du progrès social, en particulier, comme sous la IIIe République, une référence à laquelle nous sommes très attachés, vous le savez, je reste personnellement fermement attaché à l'idée d'un parlement fort comme contre-pouvoir nécessaire à l'exécutif, or c'est pas trop le cas aujourd'hui, or derrière la volonté de rationaliser l'activité parlementaire hier en réduisant le sait pouvoir d'initiative et d'amendements demain limitant, peut-être le nom se cache souvent un antiparlementarisme qui n'ose pas dire son nom, comment expliquer sinon que l'on continue de réduire le temps des débats parlementaires, jugé trop lent ça réduire en même temps, les délais d'adoption de leur décrets d'application : comment de la même façon, expliquer que contraignant notre droit d'amendement pour lutter contre l'inflation législative, lorsqu'on constate que le part considérable des articles additionnels adoptés, a laissé un, ce sont d'origine gouvernementale, il est pourtant évident que le premier obstacle à la qualité du travail parlementaire et la difficulté à bénéficier au même titre que le gouvernement de l'expertise de l'administration, or les rapports des inspections générales où sont quasiment inaccessible, quand bien même nous apprenons leur existence, ça dans son dernier rapport d'activité, le Conseil d'État, constate également la faible quantité d'études d'impact annexé au projet de loi, cela ne fait que confirmer en réalité que la loi organique du 15 avril 2001 relative notamment à l'application de l'article 39 de la Constitution, à l'évidence, il obtint à bien des égards, il semble que les parlementaires soient devenus les fusibles d'un régime de gouvernance qui apparaît à la croisée des chemins, condamné à porter la responsabilité de dispositions législatives sur lesquelles ils ont de moins en moins de prise, la procédure de lait de législation en commission vise davantage à lutter contre les effets que les causes des excès du parlementarisme rationalisé, elle risque de faire les faits donc cautère sur une chambre, elle elle n'a pas vocation à être fait quand même utilisé en raison du maintien qui a été rappelé, du droit de véto des présidents de groupe, c'est une précision nécessaire : il s'agit d'éviter qu'à l'avenir une majorité sénatoriale moins respectueuses des droits des groupes minoritaires et d'opposition, que celle-ci puisse détourner cette procédure au profit d'un passage en force, l'ouverture de la possibilité d'appliquer l'examen en commission à des parties partielle du texte pose également problème, elle n'a pas été soumise à l'expérimentation et nous considérons qu'il serait peut-être plus sage, de supprimer cette faculté et ce dans un 1er temps de même les règles de publicité les plus strictes doivent être effectivement appliquées à la commission où l'essentiel des débats se tiendra dès lors que la séance publique sera réduite à un simple rôle cérémonial conformément à l'esprit de liberté qui est l'essence du groupe RDSE et donc nous sommes d'ailleurs très fiers, plusieurs amendements compter également été déposé par notre collègue Joël Labbé, qui souhaiterait que notre débat soit étendu à la question d'une meilleure association des citoyens à nos travaux législatifs, quelles que soient nos positions sur le sujet ces propositions, je tiens à le souligner : on le mérite de montrer que certaines attributions que l'on voudrait donner à la Chambre du futur sont déjà mises en oeuvre au Sénat pour résumer la position du groupe RDSE surtout cette résolution nous soutenons totalement la démarche de la modernisation de la procédure législative, mais nous restons, monsieur le président de la commission des lois, prudent sur le fond, je vous remercie de votre grande attention. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Thani Mohamed swahili. Pour la République en marche.

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, ce président de la commission des lois, chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur la proposition de résolution présentée par Monsieur le Président, Larché visant à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission, il faut des élaborer se féliciter de cette volonté partagée de modernisation du travail législatif, disons-le sans ambages, cette initiative illustre aussi la capacité réformatrice de notre institution parlementaire, en effet, s'il est dans l'esprit du temps de construire une représentation fallacieuse de notre autre assemblée à l'enfermement dans une inertie conservatrice infondées, le Sénat ne doit pas prêter le flanc aux critiques qui l'accablent et qui viennent interroger à intervalles réguliers la pertinence du bicamérisme français. Notre assemblée doit tout au contraire démontrer sa capacité à pointer empiriquement ces imperfections interne éventuelle, les mêmes qui risquerait d'entacher la crédibilité de son travail et cette proposition de résolution s'inscrit parfaitement dans cette démarche, elle permet à la conférence des présidents de décider que le droit d'amendement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou une résolution s'exercera uniquement au sein de la commission, saisie au fond, dans ce cas, cette dernière pourra accueillir les sénateurs qui n'en font pas, qui n'en sont pas membres et ces travaux seront rendus publics comment séance les amendements adoptés par la commission, saisie au fond permettront l'établissement d'un texte qui ne sera pas examiné article par article en séance mais sera l'objet d'une présentation courtes et d'explications de vote des groupes le scrutin portant sur l'ensemble du texte uniquement sans possibilité d'un amender le contenu, par ailleurs, notons aucune innovation a été introduite, permettant de n'appliquer la nouvelle procédure qu'à une partie seulement du texte, sur décision de la conférence des présidents, quant à la séance, seuls des amendements de coordination ou tendant à assurer le respect de la Constitution ou la correction d'une erreur matérielle, pourrait être présenté si nécessaire. Voilà pour l'essentiel ici, chers collègues, le diable ne se niche pas dans les détails, cette proposition de résolution nous apporte la preuve s'il en était, que la revalorisation de la procédure d'examen en commission peut s'effectuer sans nécessairement réduire les parlementaires à leur seule fonction de tribun ni tomber dans l'écueil d'une rationalisation excessive de la procédure parlementaire, plus que jamais, il apparaît opportun de poursuivre la revalorisation du rôle déjà névralgique des assemblées des commissions délibérante amorcé par la révision constitutionnelle de 2008 quant aux éventuelles levée de boucliers, on a toujours susceptible de s'ériger contre cette résolution, au motif qu'elle porterait en germe un anti-partent parlementarisme décomplexée, il me semble utile de rappeler que le travail en commission est une phase techniques d'élaboration de la loi permettant d'apprécier au préalable la fiabilité normative de textes avant de les soumettre à l'espace de confrontation politique que nous offre la séance publique les 2 phases, loin d'être antinomique, sont en fait complémentaires, ceci est d'autant plus vrai que les garanties qui ont été apportées au texte sont de nature à apaiser les débats des garde-fous ont en effet été institué ainsi chaque président de groupe disposera d'un droit de véto qu'il pourra non seulement opposé en amont, lors de la réunion de la conférence des présidents, mais également après l'adoption du texte de la Commission pour un retour à la procédure normale, mais il conviendra tout de même de veiller à la bonne application pratique de ces dispositifs, la transposition aux différentes commissions des règles de publicité applicable à la science doit être assurée sans tarder, en définitive, cher collègue, rendons justice à notre assemblée sans revêtir le déclaration d'un esprit corporatiste qui serait assurément malvenue ne vit-on pas à faire connaître la qualité du travail parlementaire qui effectué dans le mur, cette proposition de résolution proposant de pérenniser une pratique qui a fait ses preuves, va dans le bon sens, a pourtant lui notre soutien tout en restant vigilant sur les difficultés pratiques qui pourraient se faire jour ultérieurement le groupe la République en marche soutient donc ce texte. Merci monsieur le président de la parole est à madame la présidente : Éliane Assassi pour le groupe communiste républicain et citoyen et écologiste. Pour 6 minutes, chers collègues, merci madame la présidente, monsieur le président, monsieur le rapporteur, président, mes chers collègues, en 2015, une majorité très large ici au Sénat a voté l'expérimentation de ce qui était alors la procédure d'examen en commission donc expérimenter jusqu'au 30 septembre 2017 cet objectif d'affaiblissement du pouvoir législatif, car c'est bien de cela dont il s'agit, il vous faudra bien sortir un jour des faux-semblants et la mettre cet objectif connaît sans ambages par le nouveau président de la République lors de son discours de Versailles du 13 juillet dernier n'apparaissait pas encore dans toute son ampleur la volonté pourtant la de réduire la prérogative essentielle, selon nous, du Parlement, celle de débat de la loi de prendre le temps de de le faire pour que l'intervention législative ne ne relève pas du simple travail d'enregistrement d'autres combats sur les groupes sur les bancs du groupe CRCE a toujours été celui de préserver le droit à la parole et, bien entendu, celle de l'opposition, sans laquelle le mot démocratie se vide de son sens, mais aussi d'empêcher que les assemblées parlementaires dont l'exercice même et d'être le légiste la législature Patrice ne se transforme pas j'insistant Bulliard chambre d'enregistrement, alors que le débat budgétaire se termine moments essentiels de l'année parlementaire peut-on sans rougir, affirmait que les droits du Parlement où était maintenu ces dernières années, peut-on continuer à Berne et nos concitoyens et concitoyennes en leur laissant à penser que la loi de programmation des finances publiques, non seulement d'inspiration européenne mais transcription directe des directives de la Commission de Bruxelles le traité budgétaire signé par Monsieur Sarkozy, Madame Merkel et validé par François Hollande et la déclinaison de cet engrais encadrement européen, l'article 40 de la Constitution radicalisés par la LOLF aucun impact sur la réalité du pouvoir parlementaire aujourd'hui monsieur Macron veut impulser une nouvelle étape il poussent à l'accélération des débats, la réduction de la durée de la session législative à la législation en commission enfin, faisant mine de flatter le Parlement, il vante les mérites du pouvoir de contrôle des assemblées mais cette petite musique qui fut celle du comité Balladur qui rendit ses travaux sur la réforme des institutions, il y a 10 ans fait perdre de vue l'essentiel notre système démocratique qui puisse à Sousse sa source, faut-il le rappeler, dans l'élan révolutionnaire de 1789 et la force du contrat social de Rousseau ou l'esprit de loi des lois de Montesquieu, de conférer le pouvoir législatif aux représentants du peuple, votre position constante à la Constitution de 58, trouve sa source dans l'affirmation du pouvoir présidentiel face au pouvoir législatif, or depuis le constat du coup d'État permanent par François Mitterrand, la situation s'est aggravée au détriment des assemblées, l'inflation législative, la déferlante des normes européennes, mais là en technicité et réformes essentielles : la montée en puissance du Conseil constitutionnel, affaiblissent, année après année les pouvoirs, le la révision constitutionnelle de juillet 2008 a franchi un pas important en instaurant, par exemple, le, le discours du congrès de Versailles, et surtout en s'attaquant franchement au droit d'amendement, c'est depuis cette révision, que par exemple la réforme du crédit temps véritables 49 3 parlementaires a été instauré à l'Assemblée nationale depuis l'élaboration du travail législatif au Palais-Bourbon a perdu, notamment et notablement de sa substance, qualité du travail législatif grandement détériorée à telle point que jusqu'à présent, le Sénat chambre élue indirectement par un collège de moins de 170000 électeurs, faut-il le rappeler, pouvait apparaître comme gardienne d'un travail législatif sérieux et surtout plus réaliste la proposition de résolution sur laquelle nous reviendrons en détail avec l'examen des amendements tend à pérenniser à développer la procédure de législation commission nous sommes hostiles par principe à l'instauration d'une telle procédure qui éloigne de la séance publique et du débat pleinement pluraliste, l'examen des projets ou propositions de loi destinée à cette procédure par la conférence des présidents, le Sénat semble Senor guéguerre d'anticiper sur les réformes de Monsieur Macron nous estimons au contraire que le Sénat tout particulièrement, mais aussi le Parlement tout entier si la branche la branche sur laquelle il est assis en limitant, voire en barrant la route au débat démocratique, transparent, pluraliste, le texte proposé apparaît de surplus confus, avec par exemple la législation partielle en commission, nous avons noté les doutes et les États, les interrogations de monsieur le rapporteur, qui lui-même note les difficultés qu'il y aura à gérer cette procédure tant les textes sont imbriquées entre mesures techniques et politiques, nous avons donc noter tous ses doutes mais j'espère que monsieur le rapporteur en tirera toutes les conclusions au moment de s'oppose par ailleurs comment sera géré l'agenda du parle du parlementaire si des commissions qui légifère se déroule parallèlement à la séance publique vous vanter l'ouverture des commissions à l'ensemble des élus, mais selon le droit de vote, les membres de la commission, nous entendons bien monsieur rapporteur que cette dure sera limité aux textes les moins importants, mais qui décidera de cela, l'avenir le droit de véto d'un groupe à la mise en date de cette procédure que nous avons participé, avec d'autres à préserver explicitement dans le règlement de notre assemblée, et je vous rejoins Monsieur le le rapporteur sur ce sujet est une garantie réelle. Mais jusqu'à quand le pluralisme sera-t-il respecté avec la réduction envisagée du nombre de parlementaires, que deviendront les groupes d'opposition est minoritaire dans ce qui futurs cadres qui pourra exercer le droit de véto à l'avenir, en 2008, l'article 44 de la Constitution a été modifiée pour permettent l'exercice du droit d'amendement en commission ou en séance publique, mais selon le ministre des Relations chargé des relations avec le Parlement de l'époque, notre collègue monsieur Karoutchi cette modification comme il l'a indiqué, lors de la séance du 23 juin 2008 à empêcher le dépôt en séance publique, d'un amendement, déposé en commission et rejeté la révision a donc été détournés de mon sens de de son sens pour favoriser un dangereux anti-démocratique, d'autres groupes rejettera cette propres cette nouvelle procédure car, en plus, j'ai peu de doute sur le sort qui sera réservé à nos amendements. Merci, Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Hervé Marseille pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes. Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des lois, rapporteur mais chers collègues dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 44 de la Constitution prévoit que le droit d'amendement, s'exerce en séance ou en commission. Avant cette révision, comme vient de le rappeler notre collègue la présidente à ça si les tentatives de simplifier la procédure législative s'était heurté à un obstacle constitutionnel le principe reconnue à tout particulier à tout parlementaire d'exercer son droit d'amendement en séance, en 2015 avec la nouvelle rédaction de l'article 44 nous avons pu intégrer dans notre règlement une procédure d'examen en commission, cette innovation avait pour objet de n'autoriser le droit d'amendement en commission et non en séance publique, l'idée étant, cela a été rappelé de concentrer l'exercice du droit d'amendement en commission afin de réduire le temps d'examen en séance publique, cette procédure nous apparaît intéressante après avoir été mis en oeuvre à 4 reprises sur 6 textes la conférence des présidents et au-delà, chaque groupe a pu dresser le bilan de cette procédure pour ce qui est de notre groupe, nous considérons que cette procédure a bien fonctionné, nous sommes donc favorables à sa pérennisation ainsi que modification procédurale proposée par le président du Sénat, cette opinion est d'ailleurs sauf erreur de ma pas assez largement partagée sur l'ensemble des bancs de cette assemblée, c'est parce que nous croyons à cette procédure que nous souhaitons à l'avenir qu'il en sera fait une application plus large, cela a été rappelé par le président bat le recours à cette procédure est soumis à l'accord de tous les présidents de groupe en ma qualité de président d'un de ces groupes, je suis attaché à cet aspect du dispositif et en même temps j'entrevois une possible dérive de cette prérogative, il est important de rappeler que ce pouvoir des groupes s'exercer à 2 moments initialement par une opposition préalable en conférence des présidents, le recours à la procédure de législation commission est alors impossible mais un groupe aussi s'opposer à la procédure en cours de discussion et demandé le retour à la procédure normale, c'est sur ce 2ème aspect que l'on peut avoir des observations ne pourrait-il pas constituer un moyen de pression pour obtenir telle ou telle modification sous peine de retourner à la procédure normale, on aurait peut-être pu imaginer n'utiliser que le droit de véto en conférence des présidents, la réforme de notre règlement que nous examinons aujourd'hui est donc importante et nous la soutiendrons, cela ne l'empêche pas de formuler quelques observations malgré tout à caractère plus général, le président de la République a annoncé que le gouvernement allait nous soumettre dans les semaines ou mois qui viennent, un projet de réforme de la Constitution, si cette réforme devait être adoptée, il est fort probable que nous ayons besoin d'actualiser notre règlement comme cela était le cas après la révision de 2008, aurions-nous pu attendre quelques mois supplémentaires avant d'avoir un débat global sur notre règlement, d'autant que cette question du travail en commission est expressément mis en avant par le président de la République également une autre raison repus nous conduire à différer quelque peu nos débats sur le règlement ou élargir le Champ de cette proposition de règles solution je citerai un exemple ici qui va peut-être vous faire sourire ou non, c'est la disparition de l'IRFM le 1er janvier prochain attire votre attention sur le fait que si la procédure d'examen en commission n'est plus opérationnel depuis le 30 novembre dernier une autre disposition de notre règlement ne sera plus applicable au 1er janvier les retenues financières applicables aux sénateurs en cas d'absences répétées. Je rappelle que l'article 23 bis du règlement prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un même trimestres de la session ordinaire à plus de la moitié des votes solennels et réunions obligatoires de commission, la retenue est égal à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de bombes, autrement dit notre règlement fait expressément expressément référence à lire FM comme base de calcul de cette sanction et je crains donc que cela ne soit plus applicable à compter du 1er janvier alors si heureusement évidemment dans cette assemblée, la quasi-totalité de nos collègues sont eux évidemment responsable est présent en commission, comment en séance et qu'il n'a pas été utile de recourir à cette ultime degré de sanctions, il serait souhaitable, ne serait-ce que pour la crédibilité du dispositif, évidemment qu'on en tienne compte dans notre règlement adopté en 2015, voilà une petite observation mais sous réserve de ces légères, les observations et commentaires, et non sans avoir salué l'important travail réalisé par le président de la commission des lois, le groupe union Santis Union centriste soutiendra la proposition de résolution qui nous est soumis, aujourd'hui, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste et républicain et pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, nos sommes donc amenés à nous prononcer sur la proposition de résolution du président du Sénat sur l'adaptation de la procédure de législation en commission et ça pérennisation puisque nous étions en phase d'expérimentation, ceci est possible grâce à la réforme constitutionnelle de 2008, qui, comme l'a indiqué notre collègue président Marseille a été rendue possible par l'introduction dans la constitution de la précision, comme quoi le le droit d'amendement des parlementaires s'exerce en séance ou en commission et la loi organique du du du 15 avril 2009 à organiser cette nouvelle disposition constitutionnelle et sur cette base, le Sénat a expérimenté des procédures qui nous ont permis d'adopter plusieurs lois au cours des dernières années, l'expérimentation se terminait et il était donc important de pouvoir pérenniser cette disposition on pérennise la disposition que nous avons expérimenté et finalement on a introduit une nouveauté qui aient la possibilité d'examiner partiellement un texte finalement il était pas nécessaire de refaire une expérimentation puisqu'on avait déjà fait mais on introduit une innovation dont nous verrons bien si elle peut fonctionner, mais en tout état de cause, c'était bien de pouvoir aller un peu plus loin parce qu'effectivement sur un certain nombre de textes, on peut considérer qu'il y a la partie strictement politique qui mérite une un échange en séance publique et qu'une partie, quelquefois plus technique qui peut être juste observé et étudié en commission, il me semble que cette proposition a vocation à la fois à renforcer l'efficacité parlementaire puisque un certain nombre de textes qui ne mériterait pas finalement, compte tenu du contenu des dispositions de passer à la fois en commission et séances publiques avec l'examen de l'ensemble des articles et des et des amendements peut se faire plus vite, et en même temps je crois que nous devrions aussi le voir comme une une opportunité de renforcer d'initiative parlementaire parce que lorsque j'ai lu cette proposition de résolution, il m'a semblé que pour les propositions de loi d'initiative parlementaire si effectivement des présidents de groupe qui porte ses propositions décide de les inscrire dans leur niche, ils savent que ça va prendre un minimum de temps, mais si en même temps par un accord entre les différents présidents groupes un certain nombre de PPL peuvent être et examinée sur le fond, en commission, il me semble que ça peut nous permettre de porter des propositions de loi, qui peuvent être beaucoup plus longue en terme d'articles et relativement technique, donc je je vois ça comme un un moyen de renforcer l'initiative parlementaire, si nous nous y prenons bien sous sa vont saisir cette cette opportunité en même temps je, je dois dire que on peut imaginer d'autres, d'autres sujets de transposition de textes européens qui parfois sont très techniques et et finalement qui ici ne font l'objet d'aucune discussion lorsque on dit cet article, c'est juste une transposition d'une directive européenne, ça peut nous permettent de rattraper notre retard en terme de transposition de textes européens et je vois aussi ce qui se fait dans d'autres pays, une capacité de corriger très vite nous en nous nous rendons compte que notre loi ne nous est en contradiction avec les engagements conventionnels et par conséquent il il il convient rapidement de, de, de corriger quelque chose je crois que comme tout le monde ici, nous sommes très attachés au temps législatif au fait que, même si parfois il faut être rapide et et et et imaginatif, il y a aussi un risque : il faudra être vigilant au moment de la prochaine réforme constitutionnelle le temps législatif c'est remplacer l'émotion par la réflexion, et c'est aussi sécuriser les citoyens sur la loi qui s'applique et par conséquent de temps en temps, il est important de pouvoir agir rapidement nous pourrons parler des des des sécurités qui ont été mis en place sur la disposition qui nous est proposé, mais en même temps, mais, mais il est aussi important de pouvoir sur la plupart des textes assurée par le bicamérisme et par un temps législatif raisonnables que la loi ne va pas changer en quelques jours, sans débat préalable, nous ne sommes pas d'ailleurs plus mauvais que les autres grandes démocraties ont en la matière un d'autres, d'autres pays ont expérimenté aussi ce que nous sommes en train de, de mettre en place et les observations qui se de ce qui de ce qui peut se passer en Italie, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne en particulier montre que finalement, lorsque ça se met bien en place, c'est ce que j'ai, au moment des des PPM des pour DD l'opportunité que ça peut nous offrir pour pousser plus de propositions de loi d'initiative parlementaire, il y a une capacité de négociation entre les groupes parlementaires pour justement conserver un certain nombre de textes dans ces procédures, je serai le le mot Fast Track et et ça permet finalement de bonnes négociations sur le fond des textes une rapidité, une efficacité jeudi, il faudra aussi être vigilant sur ce qui peut être le défaut de cette nouvelle procédure à lobbing moins transparent, une des textes pris finalement avec un peu moins de publicité, et aussi l'inflation législative que ça peut engendrer, si nous commençons à utiliser trop souvent cette procédure, donc il faudra être vigilant, mais c'est pas parce que on aura besoin d'être vigilant, qu'il ne faut pas soutenir cette cette initiative car finalement le droit à la fois des oppositions et les droits constitutionnels qui sont tous ceux de chaque parlementaire sont respecter au mépris de ce soir à cette tribune, l'ont dit le droit de véto des groupes est essentielle pour garantir qu'il n'y aura pas de dérives

par ce biais en disant : écoutez, si telle ou telle disposition n'est pas un peu corriger mais finalement je mettrais mon véto et on passera en séance publique, donc je crois qu'au contraire, les droits de l'opposition sont renforcés si ils peuvent être, ils sont bien utilisés, il y aura une DG dans tous les cas pour montrer les clivages et les oppositions politiques qui pourront y avoir et chacun pourra déposer des amendements, donc, et puis la la la la finalité, ce que même après un passage en commission, un président de groupe pourra demander le le le le retour à la procédure normale, ce qui vraiment permet après le passage en commission de sécuriser complètement chaque groupe parlementaire si il y a des difficultés, donc je crois que les sécurités pour respecter les droits constitutionnels et les droits de l'opposition sont sont assurés avec cette proposition de résolution qui mérite donc d'être soutenu le groupe socialiste la soutiendra, tout en défendant 2 amendements un pour avoir un un droit avec un délai d'amendements plus significative et un second pour respecter un parallélisme des formes entre les propositions de loi constitutionnelle et les projets de loi constitutionnel puisqu'aujourd'hui les uns peuvent passer dans cette procédure accélérée et les autres ne le peuvent pas voilà, je répète le soutien du groupe socialiste à cette proposition, modulo les 2 amendements que nous aimerions voir adopter et salue le travail de notre rapporteur sur ce texte, je vous remercie.

Monsieur le président. Monsieur le président de la commission des lois et rapporteur mais chaque collègue. Des la réforme de son règlement de 2015, le Sénat avait mis à profit les avancées de la révision de 2008 relatives à l'exercice du droit d'amendement en instituant la procédure d'examen en commission et se pratique expérimentale jusqu'au 30 septembre 2017. Cette proposition de résolution déposée par le président Laurent l'et vise donc à pérenniser cette procédure d'examen, tout en procédant à plusieurs adaptations pour en améliorer l'efficacité. Malgré la démission donnée à cette nouvelle procédure législation commission, texte qui en font l'objet, restons voté en séance publique, même si le droit d'amendement ne ne s'exercera plus qu'en commission, l'accueil, laquelle accueillera également l'essentiel des Ainsi, il ne s'agit pas d'un mécanisme par lequel le Sénat déléguera entièrement son pouvoir législatif en quoi une commission à l'image de ce qui peut exister au Sénat italien, si le dispositif de cette nouvelle procédure est élaboré à partir de celui de la procédure d'expérimental d'examen en commission, il en diffère toutefois en innovant sur 2 points, avec en 1er lieu la posséder d'appliquer la procédure sur une partie seulement du texte en 2ème lieu la poussée de présenter dans un cadre pré-défini des amendements en séance sur les dispositions ayant fait l'objet d'un examen en commission. Concernant la décision d'engager cette procédure. La proposition de régression stipule qu'elle reviendra à la seule conférence des présidents comme dans la prison d'examen en commission. Sur proposition du président du Sénat, du président de la commission, saisie au fond du texte du président d'un groupe où 2 nouvelles demandes. Dans ce cas, le droit d'amendement, ne s'appliquera qu'en commission. Par ailleurs, la proposition de résolution indique expressément que cette procédure n'est pas applicable au projet de révision constitutionnelle au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale. S'agissant de la Poste et de s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure de législation en commission, la proposition de réduction reprend à l'identique, ce qui était prévu dans la procédure d'examen en commission, c'est-à-dire la faculté pour le gouvernement, le président la commission, saisie au fond et tout président de groupe, de s'opposer à 2 stades. D'une part, lors de la réunion de la conférence des présidents, qui statue sur la question, d'autre part, à la suite de la réunion de la commission, c'est-à-dire au vu du texte adopté par la commission de plus, la proposition de résolution permet que soit demander un retour à la posture normale sur une partie du texte seulement que celui-ci ait fait l'objet de la posture la glisse à Sion en commission dans son ensemble, ou pour certains articles concernant l'organisation de l'appuyer des travaux, la commission. La position de région précise que les règles puissent et et le débat en séance son empire applicable à la réunion de la commission, sauf disposition contraire et que le gouvernement, comme tous les sénateurs veulent y assister ainsi ces dispositions systématise l'application des règles de la puce et en séance et permet à tous les sénateurs qui lui souhaite d'assister à la Réunion, enfin, s'agissant de l'exercer droit d'amendement en séance, à la différence de la procédure d'examen en commission, la proposition de résolution autorise le dépôt de certains amendements sur les dispositions et en fait l'objet de la procédure de législation en commission ceci concerne de la même manière, le coeur d'application de la procédure à l'ensemble d'un texte ou à une partie seulement d'un texte. Seront ainsi sans recevoir les arguments visant à assurer le respect de la Constitution, a opéré une coordination avec les textes en vigueur ou en cours d'examen ou avec le texte en discussion, enfin, a procédé à la correction d'une erreur matérielle, mes chers collègues, cette procédure simplifiée de l'eau permettent d'alléger la science publique de discussion secondaire et par là même de gagner du temps en outre grâce à l'instauration de garde-fou cette procédure restera l'exception et non la règle ainsi chaque président de groupe disposera d'un droit de véto qui pourrait opposer initialement lors de la réunion des questions et président mais également après l'adoption du texte, la Commission selon la nouvelle procédure si l'un des dépliant du groupe souhaite le retour après normal poursuit les travaux ce double véto est de nature à rassurer tout le monde, ainsi le groupe des Indes, pendant votre, cette proposition de résolution. La parole est à présent à Madame Sophie Primas pour les républicains. Et pour 15 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour des raisons circonstancielles, la commission des affaires n'a pas eu l'occasion d'expérimenter la législation en commission, selon la formule retenue entre 2015 et 2017, je sais que Jean-Claude Lenoir, mon prédécesseur l'avait néanmoins envisagé favorablement le président Philippe Bas, vient de rappeler que c'est la réussite de cette expérience et je tiens à dire d'emblée que le groupe Les Républicains votera avec enthousiasme la proposition de résolution proposée par le président Larché

trop fréquemment entre l'examen en commission et l'examen en séance publique les mêmes amendements sont bien souvent examiner 3 fois lors de la réunion en commission pour élaborer le texte lors de la réunion d'examen des amendements de séance et enfin lors de la séance publique elle-même d'une certaine manière, en déposant héros posant ces amendements, nous tentons notre chance mais chers collègues à chaque stade de la procédure ces redondances allonge débats parfois inutilement le temps ainsi gagné nous permettrait d'approfondir, d'autres débats que parfois nous devons escamoté photo de temps, mais cette procédure aura aussi pour effet de valoriser notre travail législatif en commission, elle permettra de rendre publique une partie de ce travail, elle nous permettra un dialogue Direct et vivant avec le gouvernement et elle rendra sa solennité à la séance publique qui pourra davantage se concentrer sur les textes que nous jugerons collectivement comme plus important d'un point de vue politique car nous n'avons aucune inquiétude à nourrir sur d'éventuelles restrictions de droits d'expression parlementaire, personne ne pourra imposer qu'un texte soit discuté selon cette procédure, puisque cela a été dit plusieurs fois, le gouvernement, la commission concernée au fond et surtout les groupes politiques pourront s'opposer à sa mise en oeuvre, il sera également possible de revenir à la procédure ordinaire, même lorsque la législation commission aura été engagée sur un texte, il n'est en effet pas toujours possible d'anticiper la teneur d'un débat sur un projet de loi son caractère plus ou moins intense ou plus ou moins conflictuelle, prévoir ce retour à la procédure normale et donc une disposition extrêmement sage et, quoique de plus simple que de le faire après la réunion de commission qui aura permis de comprendre qu'une séance publique de pleine exercice est nécessaire dans son rapport le président Philippe Bas précise bien que cette procédure a vocation à demeurer exceptionnel, lorsque le président, rapporteur de la commission des lois, m'a entendu, on est en audition, je lui ai fait part de ma principale remarque que la législation en commission ne soit pas une séance publique en modèle réduit, mais une vraie séance de commission, la proposition de résolution prévoit en effet que les règles de publicité et de débats en séance sont applicables à la réunion de la commission, sauf disposition contraire je pense en effet que les règles du débat doivent s'apparenter davantage à celle du débat en commission et à celle de la séance publique le débat en commission autorise des souplesses, des prises de parole multiple des durées d'intervention à la discrétion du président et non pas fixe parfois des retours en arrière s'apparentant à des seconde délibération qui permettent la vitalité, la spontanéité du débat pour parler clair, nous avons commission des débats sans papiers préparés d'avance, je vous dis à 10 en en lisant ou notre coeur, notre expérience et notre volonté s'exprime plus spontanément, c'est pourquoi j'avais exprimé une préférence pour que les règles du débat soit inspirée par celle de la scission sur ce point, la commission des lois, à mon sens la bonne réponse, ne pas importer ce que Philippe Bas appelle le formalisme, l'apparat et la rigidité de la séance publique selon à rythme ternaire que nous apprécions tous le plus simple et comme le dit la commission des lois d'appliquer les règles de la séance, a-t-il supplétifs comme un recours pour un débat dans la conduite deviendrait difficile la réussite de cette procédure dépendra également de la pratique qui sera retenu sur ce point, je le lui ai dit : je pense qu'il sera difficile de partager les textes entre partis purement technique et d'autres partis que l'on pourrait qualifier de plus sensible qu'il conviendrait de laisser aux doubles examens de la commission de la séance publique je pense que le partage reposera sur des critères qui resteront chers collègues un peu subjectif certaines parties en apparence technique pourrait se révéler en réalité plus sensible qu'au départ, d'autre part, si la commission a été amené à examiner les différentes parties dans la même journée, la demi-journée, il sera sans doute difficile de faire comprendre que la présence du gouvernement ainsi que la publicité des travaux sont réservés aux parties plus techniques, donc les peut-être les moins importantes du texte, je considère par ailleurs que le maintien de la tradition sénatoriales de laisser le gouvernement en dehors des séances législative à huis clos et souhaitables, ce n'est pas une question de principe, mais d'efficacité cette présence pourrait être source également de redondance, de redondance, j'ai donc tendance à penser que nous privilégierons l'examen des textes entiers, nous expérimentons tout ça relativement court, car il est peu probable que nos collègues souhaiteront siéger en commission plusieurs jours et plusieurs nuits sur le même texte ou de textes dont on peut penser qu'ils seront relativement consensuel, suscitant relativement peu d'amendements et peu d'affrontements, peu de débat en tout cas, ce qui n'empêchera pas un débat vivant, tels par exemple les projet de ratification d'ordonnances lorsque le Sénat aura donné son accord à la Libye, liquidation, la commission des des lois évoque aussi des textes en fin de navette en 2ème lecture notamment le texte voté en commission selon cette procédure, fera l'objet d'un débat simplifié en séance publique je souhaite insister sur un point : il sera nécessaire d'appliquer très gros rigoureusement les règles de receveur recevabilité des amendements de séance, je vous rappelle que 3 cas seulement sont prévus pour amender un texte en séance publique le respect de la Constitution, la coordination ou la rectification d'erreur matérielle, il faudra éviter que ne soient rappelés des débats de fond de façon détournée, cela a pu arriver par le passé à l'Assemblée nationale sur des articles pourtant fermée par des étapes antérieures de la discussion, enfin, une question me paraît devoir se poser, celle de la concomitance de la législation en commission avec d'autres débats, il a été d'ailleurs posée par Madame Assassi Madame la présidente assassiné l'actuelle procédure d'examen en commission est exclusive de la séance publique mais autorise d'autres réunions de commissions, comme il est probable que l'application de la législation commission appliquera de siéger plus longuement aux commissions, cela pourrait conduire à reléguer les réunions de certaines commissions et même la séance publique en soirée et la nuit, alors même que ces instances n'aurait pas pu siéger la journée à première vue, cela ne paraît pas souhaitable mais d'un autre côté, la législation en commission étant ouverte à tous les sénateurs, le problème de l'éventuelle simultanéité des réunions se posera pour certains de nos collègues, il faudra donc bien organiser le planning en conférence des présidents pour conclure j'aimerais souligner que cette nouvelle procédure est une Pierre de plus dans l'édifice de réformes que nous avons entamé en mars 2015 et qui se poursuivra bien sûr avec la réforme, la révision constitutionnelle que souhaite le président de la République et à laquelle le Sénat travaillent déjà dans un esprit je n'appellerai pas constructif mais novateur en tous les cas dans notre République, l'Assemblée nationale n'a plus beaucoup de marge de manoeuvre, puisque le gouvernement le lui en laisse guère, elle doit toujours approuvé l'essentiel des projets de loi, cela n'a rien d'indigne, c'est la logique majoritaire, qui est un des fondements de la solidité des institutions voulue par le général de Gaulle et depuis 1958 rarement les Français en ont eu à s'en plaindre, mais la contrepartie est que nos collègues députés ont de plus en plus tendance à multiplier les détails dans les textes, faute de pouvoir peser sur les sujets de fond nous sénateurs devant avoir une ambition plus large, nous, fustigeant l'inflation normative, nous devons donc faire la chasse aux lois obèses aux lois bavardes aux lois protéiforme et recentrer les textes sur quelques prescriptions nécessaires, comme nous l'avons commencé sous l'impulsion des présidents Larché bah, nous devons appliquer strictement les risques il recevabilité traquer les dispositions sans lien avec les tests, les textes en discussion et celles ne relevant pas du domaine de la loi, nous devons aussi nous discipliner chers collègues dans l'usage de notre doit d'amendements, cesser de redéposer sans cesse les mêmes abonnements car la législation délégué n'aura qu'un effet restera sur le débat de ce point de vue, bref, pour éviter que ne tombent, les bras de grand législateur sur le regarder quel nous sommes constamment dans cet hémicycle le Sénat se doit d'être et de demeurer le gardien exigeant de la qualité de la loi, je vous remercie. La discussion générale est Close, nous passons à la discussion du texte de la Commission. Et nous arrivons à un article additionnel avant l'article unique, un endroit, un amendement rectifier défendue par monsieur Boucher. monsieur Boucher. être candidat pour cet amendement de considérer qu'il est défendu. Merci, cher collègue. Quel est l'avis de la commission. Favorable défavorables. Merci mais ce président. Je n'ai donc on voit l'amendement rectifier bis qui a accueilli un avis défavorable de la commission qui est pour. qui est pour. Il n'est pas adoptée. Toujours avant l'article unique, un amendement 13 rectifier défendue par monsieur Collin tout aussi brillamment. Merci monsieur le Merci monsieur le président, chers collègues, le 3ème alinéa de l'article 40 de la Constitution dispose que la discussion : un service public en première lecture ne peut intervenir dans la première assemblée saisie qu'à l'expiration de mener de 6 semaines après son départ dans la 2ème assemblée saisie, il est de 4 semaines au moins après sa transmission cette règle vise à garantir que les parlementaires disposent d'un délai raisonnable pour examiner chaque projet ou proposition de loi va sa discussion assez délais s'ajoute celui prévu par le règlement de notre assemblée, devenu absolument nécessaire depuis la réforme de 2008 et la règle de l'examen du texte de la Commission 16 public, il vise à garantir cette fois que les sénateurs disposent de 22 raisonnable d'examen entre la modification du texte en commission et son examen séance publique, l'article 28 du règlement fixe ce délai à 2 semaines, qui peut être réduit à une semaine en cas de décision favorable de la conférence des présidents lorsque quand c'est souvent le cas au Sénat, le texte, famille et 13000 depuis l'Assemblée nationale et que c'était c'est Psion est impliqué, cela signifie que le rapporteur dispose de 3 semaines pour proposer sa version du texte, tandis que les autres sénateurs, s'ils veulent modifier le texte commission ne dispose en réalité que de séjour entre mercredi, date de la réunion de la commission et la date limite de dépôt souvent arrêter le lundi suivant, j'espère que tout le monde a suivi, il s'agit de fenêtre d'opportunité extrêmement réduite dans chacun mesure ici les implications du point de vue de la qualité des amendements déposés, a fortiori lorsqu'on ne dispose pas de l'appui des administrateurs en commission, c'est pourquoi nous proposons que dans les cas particuliers de la procédure de législation commission déception de réduction du délai de 2 semaines, à une semaine soit rendu impossibles afin de nous permettre un examen sereine dép modification introduite par le rapporteur et si besoin demander le retour à la procédure normale, cette solution a l'Avantage d'améliorer la qualité du travail législatif sans croire de pour cela, le temps des discussions en commission et séances publiques et bénéficierait talons Membre du des groupes minoritaires et d'opposition, ceux du groupe majoritaire, je vous remercie d'adopter, bien sûr, c'est excellent amendement. Merci, chers collègues, je vais demander l'avis à la Commission. parce que nous rentrons avec la législation en commission dans un régime de souplesse, la conférence des présidents, prendra une décision, mais vous savez bien que dans le parcours ordinaire d'un texte de loi, les délais sont selon qu'il s'agisse de la première ou de la seconde assemblée saisie de 6 semaines 4 semaines mais quand eux la procédure dite accélérée est appliquée ces délais et je crois que la meilleure 40 que nous aurons le temps de procéder à un travail de fond sur ces textes qui, on peut le penser, ne seront pas les plus complexes dont nous ayons à délibérer, je crois qu'il faut faire confiance à la conférence des présidents en se disant que de toute façon le droit de véto de chaque président de groupe et la garantie absolue et radicale que ce débat en commission ouverte se déroulera en laissant à tous nos collègues, le temps nécessaire pour que le travail soit un travail de qualité, c'est la raison pour laquelle je préférerais que vous retiriez votre amendement au bénéfice de cette explication un peu empirique, sinon, je dois confirmer l'avis défavorable de notre commission des lois. Merci, monsieur le rapporteur, chers collègues, merci, il est retiré. Toujours avant l'article unique, nous sommes saisis de 2 amendements identiques, le 15 rectifier bis défendue par monsieur Artano. Merci monsieur le président, nous nous apprêtons à discuter le texte visant à simplifier notre procédure législative au Sénat en favorisant le débat en commission élargie tout on amoindrit sans le poids de la séance publique cette dernière sera réduite à sa plus simple expression, à la correction des erreurs matérielles et aux amendements de coordination, le rapport est fait de rendre notre travail encore plus difficilement compréhensible pour nos concitoyens, à moins évidemment qu'on établisse un certain formalisme en commission et que l'on accepte enfin que celle-ci soit filmée et diffusée en Direct, au même titre que la séance publique. Cela d'ailleurs déjà à l'Assemblée nationale, ainsi, nous proposons un amendement qui va dans le sens du rapprochement avec nos concitoyens, afin de les inciter à participer à nos travaux en émettant des avis et des propositions sur une plateforme dédiée sur le site du Sénat, il existe déjà des espaces participatifs sur notre site internet, il conviendrait toutefois dans l'améliorer l'ergonomie et surtout de publier les résultats de ces consultations dans nos rapports afin de pouvoir en débattre en hémicycle. Surtout, cet amendement est un message pour nos concitoyens, nous disons que nous souhaitons travailler avec eux et nous les écoutons et que nous sommes à leur disposition pour leur expliquer ne les décisions que nous prenons. Le Sénat montrerait en adoptant cet amendement, sa capacité à adapter son fonctionnement aux nouvelles attentes des citoyens qui ne se limite pas à l'accélération de la procédure législative, merci monsieur le président. Qui sont en discussion commune, ils sont en discussion commune tout à l'heure, j'ai dit par erreur qu'ils étaient identiques, ils sont en discussion commune hé ben votre présenté successivement avant la l'avis de la commission. Merci donc c'est l'amendement numéro 16 articles additionnels, il s'agit d'un amendement de repli très similaire au précédent dans cet amendement, l'espace participatif est ouvert seulement à la demande du rapporteur, nous avons également enlever la mention d'une publication dans le rapport des propositions soumises par nos concitoyens, on l'état il s'apparente à la pratique actuelle de la haute assemblée, il s'agit donc uniquement de consacrer cette pratique dans notre règlement, sans que cela puisse perturber nos modes actuels de fonctionnement. nous vous disons que nous envoyons à nos concitoyens est important dans le cas où le taurillon le Sénat simplifie sa procédure législative, tout en incitant les citoyens à participer à ces travaux, merci. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. Monsieur le président, des lois recourent d'ailleurs régulièrement, ça a été le cas pour la réforme de la justice et donc pas sur un sujet secondaire mais mon cher collègue, nous n'avons pas besoin de voter cet amendement pour faire vivre des espaces participatifs, en revanche, si nous le votions nous commettrions une inconstitutionnalité, ce qui serait regrettable pour notre haute assemblée car vos amendements prévoit aussi. Que dès amendements pourraient être rédigé. Dans le cas de ces espaces participatifs et qui devrait être ensuite discuté par notre assemblée, mais ça c'est inconstitutionnel, nos concitoyens n'ont pas le droit d'amendement, c'est le principe représentatif nous parlementaires nous représentons la nation et nous avons avec le gouvernement, le monopole de l'initiative législative, on peut faire évoluer cette doctrine, mais à ce moment-là il faudra réviser la Constitution, précisément, nous avons la chance d'avoir un exercice de révision constitutionnelle qui a des chances de de s'ouvrir dans un proche avenir, profitez-en, à ce moment-là, pour faire progresser vos idées. je, je rejoins pas les les conclusions du du rapporteur appartiendront on va, on va donner justement en commission rapporteur un pouvoir de fait bien plus important, je pense que cet espace participatif doit être l'occasion justement pour lui d'avoir une vision plus plus général des différentes propositions qui sont faites pour améliorer la loi parce que comment ça se passe jusqu'à présent, on a tous ici et là et des propositions d'amendement qui nous viennent de gens proches de gens bienveillants qui nous rédige amendements, c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec 3, 4, 5 fois le même amendement déposé en en en séance et donc cet espace participatif en fait d'une certaine manière, il passe par les parlementaires en Direct et par Mail l'espace participatif, en plus d'offrir à des citoyens non organiser un espace pour faire aussi des propositions permettraient rapporteur d'avoir une vision plus plus général de tout ça, évidemment, mais c'est pas dans c'est pas dans l'amendement c'est pas dans l'amendement de donner un pouvoir d'amendement à cet espace participatif, tout cela reste totalement sous le contrôle du rapporteur et simplement et notamment dans l'amendement repris, on dit juste : il fera un rapport de ce qui a été dit dans l'espace participatif, mais ça va nourrir et vu parce qu'on discute ce matin qui est bien d'avoir un travail en commission, plus important, je crois que ça serait oeuvre utile de donner cet outil complémentaire au rapporteur, qui du coup pourrait mieux équilibrer son rapport et ses propositions d'amendement, mais en tout cas c'est pas anticonstitutionnel, il y a pas marqué dans l'amendement qu'on donne un droit d'amendement à l'espace participatif.

était à une technique que nous utilisons aussi souvent ou en tout cas que nous avons utilisé en particulier à la commission des lois à titre personnel, je l'avais utilisé lorsque nous avons examiné la loi dite sapin 2 petits personnages l'inutilisés également lorsque nous avons discuté de la PPL sur l'efficacité de la justice, nous avons fait un espace participatif et je peux vous assurer que nous avons analysé lui tout ce qui nous était relaté sur cet espace participatif je souhaite personnellement que, effectivement, nos concitoyens par ce biais, signe ici plus au débat parlementaire et en tout cas, il participe plus, je dois vous dire que dans les expériences que j'ai tenté, la déception est quand même réelle car nous avons eu peu de participation sur Sears pas qui était précisément fait pour qu'il y en ait. Je n'ai aux voix l'amendement 15 rectifier bis qui a recueilli un avis défavorable de la commission qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour le 16 rectifier bis même voilà merci. Nous passons à l'article unique et Monsieur Philippe Adnot a demandé la parole. Merci monsieur le président, mes chers collègues, je n'ai pas pris la parole dans la discussion générale je ne reprendrai pas la parole pour expliquer mon vote donc ce que je vais dire maintenant sur l'article servira pour l'ensemble, je ne vais pas m'opposer à ce texte, alors même que je considère qu'il est une remise en cause grave du pouvoir des parlementaires, je vais pas m'opposer à ce texte parce que il y a eu des garde-fous parce qu'il y a la capacité pour les commissions et pour les groupes de dire Stop, on ne veut pas que ce texte passe sous cette formule, c'est donc une garantie, mais il faut que vous soyez tous conscients que nous allons instituer un système où un parlementaire n'aura plus le droit de vote sur un texte qui leur a proposé. Puisque à parlementaire qui n'est pas membre de la commission peut venir défendre son amendement devant la commission, mais ne peut pas participer au vote, donc ce qui veut dire que, ne pouvant pas participer au vote dans la commission ne pouvant pas participer au vote dans la séance publique puisqu'on n'examinera pas les amendements en séance publique les parlementaires que nous sommes allons voter un texte qui va nous diminuer notre pouvoir réel tant que ça restera sur des textes limité d'accord. Mais si un jour la dérive existe pour des raisons qu'on peut imaginer, je pense que nous aurons procédé là aujourd'hui à une remise en cause grave du pouvoir de chacun d'entre nous, il aurait fallu permettrait aux parlementaires qui vient défendre un texte devant la commission qu'il est aussi le droit de vote, devant cette commission parce que sinon ça veut dire que plus jamais il ne peut s'exprimer, alors les groupes pourront toujours dire mais dans la commission, nous avons des parlementaires qui peuvent relayer, sauf que c'est le tropisme d'une commission qui s'exercera pour décider et ça n'est plus le pouvoir de l'ensemble des parlementaires j'attirer votre attention sur cette remise en cause, que je considère assez grave. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur, ce président.

je reconnais bien volontiers que dans nos débats à l'intérieur de l'hémicycle. Des amendements qui ne font pas l'objet d'un avis favorable de la commission peuvent être adoptés quand l'un ou l'une d'entre vous trouve les accents de conviction nécessaire et. Réussi à persuader un certain nombre de collègues bienveillant de participer à ce moment-là à la séance, votre serve à Sion s'aspirent de votre expérience, vous qui n'êtes pas rattaché à un groupe politique, mais il peut y avoir une autre manière de voir les choses, la régulation des travaux de nos assemblées se fait tout de même beaucoup avec une majorité et une opposition. Et le rôle des groupes politiques et très important, même si chacun est libre de ne pas y y appartenir et de ce point de vue, il y a quand même une valeur démocratique aussi au à l'affirmation d'une majorité et je dois vous dire : vous parlez comme un collègue. Indépendant et moi je vous réponds comme un président de commission, chacun est bien dans son rôle mais il y a une méthode arrivé de ressentir comme une forme d'embuscades lorsque nuitamment un amendement est adopté alors que l'hémicycle c'est soudain composé de collègues qui se trouve être en faveur de cet amendement et cela peut conduire à à des incohérences dans un texte que l'on discute, c'est la raison pour laquelle, tout en reconnaissant la valeur de votre argument, je n'ai pas souhaité dans les amendements que j'ai présentée sur ce projet de résolution lui donner de conséquences juridiques précises, j'admets que c'est pour vous une perte de chance mais je suis également sensible à ce que on ne modifie pas la cohérence et l'équilibre d'un texte en ayant réussi en fonction des circonstances d'un débat à faire adopter parfois dans une sorte d'improvisation, un amendement qui serait contraire à la position de la Commission. défendue par Damas si monsieur Ouzoulias. Seul président mais, chers collègues, nous voulons par cet amendement réaffirmer notre proposition de fonds à la procédure de législation commission à l'heure où il existe une réelle volonté politique exprimée fortement par le président de la République de réduire les pouvoirs et les droits du Parlement, il nous semble risquer de lui donner des moyens de mettre en oeuvre cette politique aux dépens de la liberté de notre haute assemblée outre notre position de fond nous relevons dans la proposition des incohérences ou des approximations qui pose, selon nous, le problème de la crédibilité du dispositif proposé, vous avez vous-même, monsieur le rapporteur, quelques interrogations sur cette disposition, vous soulevez notamment le caractère aléatoire et parfois complexes de la délimitation entre les mesures dites techniques et celle plus politique, la question de la recevabilité d'amendements sur les dispositions examiné en séance publique n'est par exemple pas résolu de manière satisfaisante, comme nous le pensons, pour justifier une éventuelle extension de la législation commission vous ouvrez à l'ensemble des sénatrices et sénateurs, la réunion de la commission saisie mais seuls les membres de cette commission ont le droit de vote peut-on considérer que le droit d'amendement de l'ensemble des sénatrices et sénateurs et respecté, alors que ce droit de vote n'est pas reconnu la question mérite d'être débattue, autre interrogation : l'arbitraire de l'organisation des débats de commission sera laissée à la discrétion de leur président ou présidente, ce sera une législation à Jean Mitry variable sans droit préétabli pour l'opposition, en particulier le respect du pluralisme, alors que les petits groupes ne dispose que d'un ou 2 membres en commission et aussi loin d'être assurée, enfin, nous avons obtenu le rétablissement explicite du droit de véto pour les présidents de groupe, c'est une garantie, mais pour aujourd'hui, que se passera-t-il demain par exemple du fait de la réduction du nombre de parlementaires et du maintien d'un mode de scrutin imparfait, si l'opposition n'est plus représenté sous forme de groupes et dans la situation de recomposition politique c'est pas une hypothèse absolument aberrante toutes ces objections, nous amène à proposer la suppression de ce projet, procédures de législation en commission, je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, oui, vous venez de rappeler la la la la la position de votre groupe, dont je ne conteste d'ailleurs pas la la cohérence pour autant au cours de ces débats et au cours de la présentation dans la discussion générale, il a été clairement indiqué quels étaient les intérêts de de de cette procédure qui, encore une fois n'est pas appelé à remplacer, dans une large mesure la procédure normale et puis surtout, il y a, c'était dément que personne ne doit oublier dans l'hémicycle, c'est qu'à tout moment, vous pouvez y mettre fin, un président de groupe et y mettre fin, tout est dit, lorsqu'on a lorsqu'on a dit cela, alors votre position et cohérente, c'est pas celle de de la commission puisque votre amendement, reviendrait à supprimer totalement le texte que nous examinons donc c'est évidemment un avis défavorable à rendu la commission. Merci monsieur le président je mets donc on voit l'amendement 19 qui a recueilli un avis défavorable de la commission qui est pour.

le Champ d'application de la peine, c'est un peu leur la part sans nom barbare est une question essentielle : fallait-il limiter son application à certaines petit peu de texte dès lors que le droit de véto des présidents de groupe était consacré dans sa décision du 11 juin 2015 le Conseil constitutionnel a considéré que certaines taxes ne pouvait se voir appliquer cette procédure en raison de leur soumission à des dispositions particulières du règlement du projet de loi constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la Sécurité sociale, cela revienne finalement à reconnaître qu'il pourrait exister des dérives dans l'application de cette procédure, dès lors qu'aucun obstacle juridique nous empêche de réduire un peu plus le Champ d'application de la PLC au-delà des limites fixées par le Conseil constitutionnel le cas particulier des résolutions mérite notamment d'être puisqu'elle ne constitue pas à proprement parler des dispositions législatives ou alors le sens de cet amendement que je propose, bien sûr, la note. Monsieur le président le la commission a délibéré de cet amendement et a émis un avis. Défavorable, là encore, je reprends ce que disait le président Pinel instant le droit de véto des groupes empêchera une application qui pourrait être jugée politiquement inopportune, c'est la raison pour laquelle notre avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur.

Oui, monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, la proposition de résolution prévoit qu'il ne peut être recouru à la procédure de 10 stations commission pour le projet de révision constitutionnelle, les projets de loi de financer et des projets de loi de financement de la Sécurité sociale, cela s'explique par le fait que ces 3 types de projets de loi donne Paluel, élaboration d'un texte en commission toutefois pour un parallélisme des formes entre les propositions de loi constitutionnelle et les projets de loi constitutionnelle, nous proposons d'élargir cette exception au proposition de loi constitutionnelle, même si nous nous reconnaissons que pratiquement, il est probable qu'un président de groupe, qui souhaite inscrire une proposition de loi constitutionnelle souhaitera aussi, que ça soit discuté en séance publique,

défendue mais rappelle que notre endettement vouloir mettre sur le même plan les projets et les propositions de loi constitutionnel procède de la volonté de défendre les droits du Parlement que j'exprimais tout à l'heure dans la discussion générale, le rééquilibrage institutionnel entre le Parlement et l'exécutif nécessite en 1er lieu que les parlementaires refusent d'intérioriser les limites de la portée de leur action imagine autant quelque gouvernement que ce soit, reconnaîtra la valeur supérieure d'une proposition de loi sur un projet de loi imaginables cette résistance se passe par la reconnaissance des mêmes garanties procédurales loi constitutionnelles qu'elle soit d'origine gouvernementale ou qu'elles soient d'origine parlementaire, c'est le sens de cet amendement que je vous propose bien sûr notre. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. Monsieur le président, je dois vous dire que j'ai de la sympathie pour c'est vous amendements et que je me suis fait un peu violent pour les rejeter, mais je les fais par devoir parce que il y a une. Cohérence dans votre approche, c'est de dire, puisque les projets de révision constitutionnelle ne peuvent pas faire l'objet de cette procédure dont nous parlons, alors pourquoi les propositions de révision constitutionnelle pourrait en faire partie et je trouve que la question est légitime, d'autant plus que la Constitution, c'est tout de même très important, personne ne dira le contraire, mais en fait il y a une raison oui et cette raison elle est assez simple, c'est que dans un projet venant du gouvernement pour réviser la Constitution, la commission de l'adopte pas de texte de la Commission, on vient en séance avec le texte du gouvernement et donc ça rend absolument impossible le l'application de la procédure de législation comme ici, on ne peut pas le la concevoir, dans ce contexte-là, en revanche, dans les propositions qui émanent de parlementaires de révision constitutionnelle, il y a bien l'établissement par la commission d'un texte de la Commission, il y a ce moment-là la procédure dont nous parlons, pourrait se concevoir, mais elle pourrait se concevoir juridiquement à l'État inconcevable, politiquement, cela va de soi, mais si nous admettons de faire une entorse à la règle générale que je rappelais seules sont exclues de la procédure législation commission les textes qui ne font pas l'objet d'un texte de la Commission, on doit rejeter ces amendements et vous verrez tout à l'heure ça une petite importance quand même parce que viendra la question des lois organiques qui sont supposés très importante de, nous avons vu à l'instant, la question des résolutions sur le règlement et si on se met au fond à décider qui il y a, en fonction de l'importance des textes, des règles qui doivent être posées dans notre règlement, on va pas en sortir, je crois que il faut là encore se dire que la seule vraie garantie les politique c'est le véto qui imaginerait qu'on aille réviser la Constitution en faisant de la législation en commission est ce qu'il y a un seul d'entre nous qui imagine ça, moi je ne le crois pas, donc je vous demande de bien vouloir rejeter cet amendement qui m'est sympathique et qui est inspirée par une vision exacte de l'importance des textes constitutionnels dans nos travaux, mais qui nous mettrait en face d'un problème de cohérence avec beaucoup d'autres exclusion possible du Champ d'application de la procédure de législation en commission. Merci, monsieur le rapporteur monsieur Guillaume le président Guillaume pour explication de vote. Oui, monsieur le président, Monsieur le président de la commission votre brillante argumentation n'amène à penser que vous auriez dû dire : j'ai donné un avis favorable à l'amendement qui est proposé dans la logique a donc peut-être aller à, encore, encore un effort, Monsieur le président, les parce que quand même une réviser la Constitution, ce n'est pas rien, ce n'est pas une exception, comme les autres, vous dites : il peut y avoir beaucoup de d'exception évidemment et puis beaucoup d'exceptions, mais là nous parlons de révision constitutionnelle, je pense qu'on peut tous s'accorder dans cet hémicycle pour dire: il peut y avoir d'autres d'exception que la conférence des présidents et souveraine que le véto d'un président de groupe peut faire tout cela, c'est pour ça que tourne favorable votre texte, mais même dans ce texte de façon très forte et symbolique que il ne peut pas être débattue dans cette procédure, tout ce qui touche à la constitution, il me semble que c'est un un meilleur verrou que la conférence des présidents et que l'on peut le véto d'un président de groupe, c'est tout simplement le Sénat qui dit : cette procédure est du pour séduire, qui va dans le bon sens qui accélère, mais franchement, en tout état de cause, quelles que puissent être les autres dérogations celle-ci révision constitutionnelle n'entre pas dans le Champ de ce texte. Merci, cher collègue Monsieur qu'on a, explications de vote. Cet amendement, monsieur le président, vous l'avez enterré sous les fleurs, mais je suis persuadé que cette assemblée a été sensible à cette brillante argumentation et que bien entendu nous allons adopter cet amendement, je vous remercie. Merci, cher collègue, je n'ai donc on voit ces 2 amendements identiques qui ont fait l'objet d'un avis défavorable mais sympathique du rapporteur qui est pour. qui est pour. Nous allons recompter, qui est pour l'amendement des amendements.

Qui est contre

Collin. Le président. Mais, chers collègues n'y voyait pas d'acharnement de ma part. Je souhaitais simplement souligner que notre droit constitutionnel réserve également l'organique des garanties procédurales spécifiques Alien avaient leur place dans la hiérarchie des normes. normes. Dès lors, permettre de les soumettre à une procédure législative si confidentiel je n'ignore pas que l'organique a déjà été adopté selon cette procédure, il s'agissait de démarche dématérialisé, le Journal officiel, sujet sensible s'il a peu peu temps d'une expérience et si précisément consensuelle tirer la conclusion que cette procédure sera utile en matière organique, je ne le crois pas, je vous remercie de votre attention. Alors là, mon cher collègue, c'est différent. Non, parce que, parce que figurez-vous. Que sur 4 lois adoptées en application de cette procédure, il y en a 2 qui était organique. Notamment la célèbre loi sur la dématérialisation du Journal officiel, parce qu'il peut se trouver qu'il y a des dispositions de loi organique qui n'est pas une importance universelle, ni même une importance cosmique. Mais qui soient à leur place technique. L'objet de cette procédure, donc là pour le coup, c'est pas comme pour la constitution, tout dans la Constitution est très important et dans les lois organiques, il y a des choses qui sont qui sont fondamentales et d'autres qui sont plus techniques et donc si, peut-être que vous accepteriez au bénéfice de cette explication de retirer votre votre amendement.

monsieur le président, Michel collègues l'alinéa 8 de la proposition de résolution ouvrant la possibilité de recourir à la procédure de liquidation de commission pour des parties de texte également nous nous opposons à cette possibilité pour diverses raisons en 1er lieu cette faculté n'a pas été expérimenté dans le Tarn imparti par la précédente résolution compte tenu des nombreux problèmes techniques que la mise en oeuvre est susceptible de comporter cette expérimentation aurait pourtant été me semble-t-il, très utile à l'heure où nous critiquons des loi portant diverses dispositions en matière de bien connus qui ne sont que des agrégats de dispositions disparates poursuivant plusieurs objectifs parfois très éloignées, il est à craindre que ce saucissonnage parce on est moins l'expression cette fragmentation de l'examen des textes selon différentes procédures aggraver cette tendance à un salmigondis à la matière, le Parlement n'a d'ailleurs pas de leçon à recevoir du gouvernement, comme l'a relevé, fort justement, le président de l'Arche et 5ème des amendements un article additionnel sont en réalité d'origine gouvernementale, je crois que l'amélioration de la qualité, la loi passera par une plus grande cohérence de l'ensemble des dispositions intégrer un même texte au service de nombres d'objectifs resterait et elle n'est pas l'effet escompté de l'application partielle de l'PLC, c'est en fait l'ouverture de cette possibilité avec nos inquiétudes de voir cette procédure utilisée de manière plus fréquentes qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, soit 4 fois en 2 ans, vous l'avez rappelé on planifie imaginer que des dispositions jugées consensuel soient identifiées dans chaque texte soumis au Parlement, mais si les propositions de recours, partie à la procédure se multiplier les présidents de groupe devraient systématiquement procéder à un examen minutieux des dispositions mêmes causes avant même leur inscription à l'ordre du jour, ce qui n'est pas souhaitable, compte tenu des déjà très restreint que j'ai évoquais plus plutôt l'appel doit demeurer une procédure exceptionnelle et appliqué à une texte dans son intégralité, c'est en tout cas, notre sentiment est le sens de cet amendement que vous avez bien sûr adopté.

une des principales innovations de cette proposition de résolution par rapport à l'expérimentation, qui s'est déroulé de mai 2015 au 30 septembre 2017 et d'autoriser une législation partielle en commission. Même le texte pourra donc être amendée pour partie en commission pour ce qui est des dispositions jugées technique par la commission, saisie au fond et pour partie en séance publique pour les dispositions jugées politique est plus fondamentale nous sommes vous l'aurait compris en total désaccord avec ce principe et Monsieur le Président, vous y comme vous, ça crée une pleine page de votre rapport, notamment la page 37 les mots complexes difficultés subjectif, sont des mots que vous utilisez pour montrer, sans le dire l'imperfection du système proposé une question clé et, bien entendu, le caractère aléatoire de la classification des articles jugés technique ou non, nous l'avons vu à l'occasion de la loi Macron ou encore de la 1ère loi travail que 18 dispositions jugées techniques peuvent être lourde de conséquences sociales ou économiques, monsieur le président, nous nous étonnons du maintien d'un dispositif qui apparemment ne vous convenait pas, il s'agit pourtant du respect d'un droit fondamental, le droit d'amendement, ce qui nécessite de prendre clairement ses responsabilités, ce que nous proposons de faire en supprimant la législation partielle de commissions. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission pour ces 2 amendements identiques. identiques. Ce président de la commission a estimé qu'un peu de souplesse ne nuirait pas en considérant que l'un dans l'autre, il arrivait tout de même que certains textes soient sécable certains textes ça Scriva en réalité, dans la tradition ancienne dès, projet de loi portant diverses dispositions d'autres social où diverses dispositions d'ordre financier ou diverses dispositions relatives à la législation du travail parmi les dispositions, il y en a qui vraiment ne pose pas de problème politique majeur qui peuvent faire l'objet d'un examen selon la procédure de législation en commission et puis d'autres qui n'ont strictement rien à voir et ne sont pas liées entre elles. Et qui elle mérite un débat très approfondi. Selon la procédure ordinaire, c'est la raison pour laquelle la Commission a estimé devoir donner un avis défavorable assez amendements.

qu'il fallait que notre Haute assemblée se gardent des voies redondantes obèse bavarde, etc je vous suis complètement dans cette, dans cette volonté mais je pense que, pour ce faire, il faut avoir une Intelligence complète de la loi et ne pas remettre à des commissions un jugement sur des aspects qu'on estimerait a priori technique, je pense que c'est au contraire en séance que nous devons, comme nous en avons les possibilités considérer que certains articles revêt relèvent du domaine réglementaire et doivent être repoussé, sinon, on estime qu'il y a finalement 2 possibilités d'examens dont un, une espèce de de commissions qui ne qui ne verrait que des choses subalternes et sur lesquels il y aura un un avis technique extrêmement, je pense qu'il faut vraiment que notre commission réfléchisse et vote cet amendement pour éviter justement les les dérives que vous avez identifiées. Merci, cher collègue, Madame Prima, explication de vote. qui deviennent des débats extrêmement sensible, alors qu'on ne s'y attendait pas et qu'on s'attendait à voter quelque chose et technique, mais le président de la commission des lois a mis des garde-fous qui permettent de revenir en arrière si jamais ça ne ça ça s'avère être sensible à la sortie de la commission, effectivement, il est possible de revenir, donc je pense que les garde-fous sont sont suffisamment fort pour qu'on puisse tenter effectivement dans des conditions extrêmement précises et de couper ce texte mais comme vous, j'ai quelques réserves, mais je pense que les conditions dans ce texte de loi sont réunis pour tenter l'expérience. Merci, cher collègue. Je mets au voix ces 2 amendements identiques avec. un avis défavorable de la commission qui est pour.

Merci monsieur chers collègues cette amendement vise à réserver un thème de discussion préalable à l'examen donne texane commission par la voix de la procédure de législation en commission aux membres de la commission, saisie au fond un fait plusieurs d'entre nous ont souligné les limites liées à la présence systématique du gouvernement lors de l'examen, commission des lois qui pourrait limiter peut-être la liberté d'expression des parlementaires soutenant notamment la majorité gouvernementale, les pratiques varient d'ailleurs entre le Sénat et l'Assemblée nationale où le gouvernement n'assistent plus régulièrement aux réunions des commissions afin d'asseoir le fait majoritaire, les travaux issus des groupes de travail, à l'Assemblée suggère d'ailleurs de systèmes systématiser cette présence dès le stade de la Commission nous considérons au contraire que cette évolution et le défaut de rendre plus opaque, les travaux parlementaires et que cela pourrait donner lieu à des réunions informelles préalables dans les couloirs, comme cela est courant Paris-t-il au Parlement européen je je ne connais pas la pratique mais il paraît que c'est comme ça, bien que le Conseil constitutionnel se soit appuyée sur la mention de la présence du gouvernement dans la sa décision relative à la dernière modification de l'antérieurement sa position, monsieur le président, n'est pas clair sur la question du caractère obligatoire de la présence du gouvernement lors des réunions de commission, nous sommes favorables à une interprétation stricte de l'article 40 44 de la Constitution, selon laquelle la présence du gouvernement n'est pas requis n'est requise par donc pour l'examen des amendements et le vote, telle est l'objet de cet excellent amendement que je vous propose d'adopter bien sûr. Merci, cher collègue, qui est de l'avis de la commission. Je crois que ce n'était pas le le de Bourg-Saint-Maurice. Monsieur le président je réponds donc à la présentation de l'amendement numéro 14 par notre. Collègue Collin. C'est important. Que nous donnions. à la séance de la commission. Se réunissant selon la procédure de la législation en commission toute la solennité nécessaire Hans aspirant des règles d'organisation de nos débats dans l'hémicycle, nous ne concevons pas. Que le débat législatif puisse se dérouler en l'absence d'un ministre dans l'hémicycle. Mais puisque nous légiférons en commission, nous devons aussi avoir la présence du ministre, cette effectivement très différent de la réunion d'une commission ordinaire, je me permets de vous rappeler d'ailleurs que si les ministres exigeait d'être présent à nos réunions de commissions, nous ne pourrions faire autrement que de lait recevoir certains s'y sont, eux, essayer et au fond, ils ont fait de même le bilan de leur participation et non pas recommencer. Mais s'agissant 2. Cet exercice tout à fait particulier, je crois que, véritablement, la séance est public, le gouvernement et là, nos débats sont filmés et on s'inspire au maximum du travail en hémicycle, c'est la raison pour laquelle, chers collègues, je pense que ce serait mieux si vous acceptiez de retirer votre amendement parce que ça me gênerait beaucoup de devoir confirmer l'avis défavorable de la commission.

Les propos du président, cet amendement a pour objet, Monsieur le Président, Michel collègues de souligner les limites pratiques à l'application de la procédure de la législation commission cette version prévoit en effet que tous les sénateurs pourront y assister, y compris les sénateurs non membres de la commission, saisie au fond, il serait nécessaire de prévoir que les réunions de la commission, saisie au fond, se déroule à des horaires différents, que les horaires habituellement réservé aux réunions des commissions permanentes, c'est-à-dire le mercredi matin afin que tous les sénateurs puissent effectivement s'ils le souhaitent y participer, il s'agit d'une limite logistique non négligeables, je vous propose d'adopter cet amendement. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. Jacques Olek la souplesse est nécessaire, bien sûr, je vous. Apporte tous les apaisements nécessaires et j'en profite parce que la question est utile pour l'ensemble de nos collègues pour vous dire mais chers collègues quand, venant d'une autre commission, que la commission qui se prononce, selon la procédure de législation commission vous participerez aux travaux de celle-ci, mercredi matin, cela aura la même valeur que si vous participiez aux travaux de votre propre commission pour le calcul de votre présence dans le travail parlementaire, donc mon cher collègue, la règle est déjà posée, nous avons eu l'occasion de l'appliquer déjà puisque nous expérimentons cette procédure depuis 3 ans, n'ayez aucune inquiétude, tout a été prévu et vous ne serez pas pénalisé de participer aux travaux d'une commission qui légifère en commission. Merci, monsieur le rapporteur, êtes-vous convaincu que je Merci l'amendement est retiré, nous passons à l'amendement 21 défendu à monsieur. Monsieur le Président, donc très vite c'est un amendement de conséquences. Merci. L'avis de la commission. L'amendement puisqu'on a rejeté un précédent amendement c'est vrai.

la version actuelle de la résolution prévoit que les règles de la séance publique sera respectée, une commission mais supprime dans le même temps, certaines dispositions qui figurait dans la version du texte, expérimenté depuis 2015, il est proposé de rétablir la mention explicite de temps de parole garantie pour défendre un amendement, ce qui permet de souligner par ailleurs les limites pratiques à l'observation exacte des règles de la séance au stade de la Commission, le sens de cet amendement propose d'adopter. Merci, Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. et d'autre part, cette règle, c'est tout l'Avantage de légiférer en commission n'a pas besoin d'être opposé à chaque orateur de manière aussi rigoureuse que pendant nos travaux en hémicycle comme quoi la législation commission permet un dialogue plus souple de s'instaurer. Merci ne rapporteur Monsieur Dantec pour explication de vote. Oui, c'est un moment extrêmement important de notre collègue Colin on on sait tous comment ça se passe en commission, on sait tous comment ça se passe quand il y a 1000 amendements à traiter qu'on est un peu à la bourre, et que on est dans la proximité du d'un lieu d'un lieu réduit et que ça se finit à la chaîne, je pense qu'au contraire, à partir du moment donne un. Mais c'est partout pareil, de toute évidence, mais, mais justement, comme ça, tout ne se passe pas comme à la commission des lois, il faut renforcer la règle, c'est plutôt un argument qui qui confirme notre proposition d'amendement non la là, je crois vraiment que si on n'a pas des règles extrêmement fermes sur ce point, on risque d'avoir des frustrations, on risque d'avoir des contentieux et donc je pense que l'abonnement de notre collègue Colin au contraire sécurise le le travail de la commission, sinon je pense qu'on va avoir quelques difficultés.

la ligne 6 de l'article 49 du règlement prévoit que j'ouvre les guillemets le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de 2 minutes et demie pour un exposé des motifs, cette disposition prévue pour la séance publique sera donc applicable à la réunion de la commission d'enquête de la procédure de législation commission vous êtes parfaitement rassuré manifester le vous êtes rassuré. Que amis chers collègues, si la réforme proposée vise à accélérer la procédure législative ne doit pas aboutir à ce que les sénateurs qui n'ont pas pu être présent commission ne puissent pas accéder à l'intégralité des débats, nos concitoyens doivent pouvoir comme cela est le cas d'un examen national se consulter le compte rendu intégral des débats le présent amendement a donc pour objet de préciser que les comptes rendus des débats en commission est intégral et non pas détaillé, je vous remercie parce que c'est un très important, je vous propose d'. Merci, cher collègue que le même et défendu par Madame Assassi. Oui, merci Monsieur le Président, c'est tout à fait le même que monsieur celui monsieur Collin, il est tout aussi important et donc je vous demande aussi de d'adopter ces amendements. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission sur les dix, rectifier les 22. Il est défavorable mais, chers collègues, il y a un compte rendu détaillé de nos travaux en commission qui va bien au-delà du compte rendu analytique de nos travaux en séance et qui je crois suffit amplement à informer le public que de la réalité des propos qui ont été tenus. Merci ce rapporteur je me vois ces 2 amendements identiques. Qui est pour. Qui est pour. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptées le passons un amendement numéro 23 défendue par Madame la Présidente Assassi. Merci Monsieur le Président, riches vers le 23 et le 24 sur le 23, nous estimons que, comme pour la séance publique le compte rendu analytique des débats en commission devra être le plus rapidement possible disponibles dans le cas de la procédure de législation en commission et en particulier de législation partiale, pour mesurer les impact potentiel sur les dispositions conserver pour le débat en séance publique et quant aux 24 c'est un amendement qui vise à faire préciser l'ordre lors de nos, d'autres de notre débat, un point qui nous semble important, bien évidemment, nous approuvons que le retour à la procédure normale puisse être demandé après l'examen d'un texte en commission sur le régime de la nouvelle procédure de législation et en particulier par un président ou une présidente de groupe, la fin de l'alinéa concernés par d'autres amendements évoque la possibilité d'une opposition de la conférence des présidents des présidents cet alors c'est une question cette opposition porte-t-elle sur le principe même du retour à la procédure normale ou sur le délai durant lequel ce retour pourra être demandé donc j'espère avoir une réponse sur ce point. Merci, cher collègue, la parole est à la Commission. Sur la moment 23 qui demande quand même compte-rendu analytique. soit. Soit ajouté, je crois que compte rendu détaillé suffit largement, et donc l'avis de la commission est défavorable et sur l'amendement 24 qui prévoit la la suppression de la possibilité pour la conférence des présidents de modifier la date butoir pour demander le retour à la procédure normale, nous avons considéré que cela rigidifie Ray inutilement les choses alors que toute garantie sont déjà apporté que ce retour à la procédure normale pourra Dender qui déraisonnable être obtenu. Merci, monsieur le rapporteur, je mets aux voix l'amendement 23 monsieur Leconte pour l'explication de vote. Oui merci monsieur le président, ne semble que si on veut effectivement sécurisé la procédure de législation en commission, faut-il mettre un minimum un maximum de garanties, je crois que cet amendement effectivement propose inscrit précisément un minimum d'exigences et de transparence et de rapidité dans la publication d'un compte rendu analytique qui peut peut-être rassurer ceux qui doutent de l'efficacité de cette procédure et pour tout le monde, ce sera de la transparence, donc je crois que ça, de ça, plus c'est plutôt ça serait plutôt de bon esprit que d'adopter cet amendement. Merci, cher collègue, je le mets donc on voit avec un avis défavorable de la commission qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient l'amendement 23 n'est pas adopté est-ce que c'est le même vote pour le 24 même vote merci, nous passons à 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune

il y a, à mon sens une rigidité trop importante des délais pour déposer des amendements dans un certain nombre de cas, et c'est un amendement vise à rétablir un droit effectif d'amendement en séance, en cas de retour à l'examen, dans l'hémicycle, parce que quand on regarde la manière dont s'est rédigé aujourd'hui on pourrait se retrouver dans des situations où en réalité nous aurions que quelques heures pour déposer des États amendements, ce qui n'est pas très très correct et et donc nous proposons de revenir automatiquement à une décision de la conférence des présidents, qui aura la sagesse à ce moment-là, de donner un délai raisonnable qui permette effectivement d'exercer un droit d'amendement qui dans certains cas, pourrait être menacée si nous n'adoptions pas cet amendement, je vous remercie.

il serait étonnant que le délai de dépôt d'amendements sera de texte en cas de retour à la procédure normale, suite à la demande du gouvernement du président de la commission d'un président de groupe ne permettent pas la réouverture du délai de dépôt d'amendements, nous estimons que le dépôt, le délai de dépôt prévu à la cyclo 3 pour l'examen en commission ne peut être conservée sous peine d'empêcher concrètement le dépôt de nouveaux amendements alors que le débat a pu évoluer durant ce délai.

nous regardent, a déclaré les lois ne sont pas de pure aux actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de réseaux. C'est mots la qualité des droits se dégrader, aggravent la sécurité juridique de nos concitoyens, Mischa collègues nous concevons qu'il faille simplifier les normes ou comme le recommande le Conseil d'État que les avants demande puisse faire le l'objet d'une évaluation en termes d'impact qu'ils proviennent du gouvernement qui proviennent du Parlement toutefois le droit d'amendement, méritent d'être préservées, alors que dans sa grande sagesse, bien connu, le Sénat parvient fréquemment, améliorer la qualité des textes soumis à son examen la haute assemblée ne doit pas devenir une chambre d'enregistrement, si la réforme proposée offre la possibilité d'un retour à la procédure normale d'examen elle ne garantit pas que les délais sont ou seront suffisants pour permettre aux sénateurs d'amender le texte et ça a été rappelé par les précédents orateurs mais dans le présent d'amendements, vous l'aurez compris vise à préciser que le délai de dépôt des amendements ne peut être inférieur à une semaine, je vous remercie, propose d'adopter cet amendement. Merci, cher collègue, je vais demander l'avis de la commission. Merci monsieur le président, nous avons émis un avis défavorable à ces 3 amendements parce qu'en réalité. Le problème est déjà réglé la conférence des présidents, quand elle décide de la mise en 9 de cette procédure. Prévoit d'une part, la date de la séance publique qui est déjà arrêté et réservé et d'autre part. Il prévoit aussi la date limite pour la présentation des amendements en séance publique, car j'ai dit tout à l'heure à la tribune d'une manière trop brève que la possibilité d'amendements, c'est quand séance publique survit par exception à la règle selon laquelle, le texte est adopté intégralement commission et qu'on y touche plus, il y a en effet plusieurs types d'amendements qui pourront être présenté des amendements pour corriger une erreur matérielle des amendements aussi pour se conformer aux exigences constitutionnelles, si par malheur le texte adopté en commission était contraire à certaines dispositions de la Constitution ou les amendements de pure coordination du coup au moment où on décide la mise en 9 de la procédure, on décide aussi d'une date limite pour les amendements que personne parmi nos collègues ne pourra ignorer, du coup, ça n'est pas nécessaire de prévoir les amendements qui viennent de nous être présentées et par ailleurs il amène une difficulté qui risque vraiment d'être lourde, c'est que si la commission s'est réunie le jeudi, supposons ensuite le président d'un des groupes disent : nous devons nous voulons rétablir la procédure normale et que l'on doive à ce moment-là, réunis à la conférence des présidents ne pourra le faire compte tenu du fait qu'on aura retenu une date pour la séance la semaine suivante, on ne pourra le faire que le vendredi, voir le samedi, ce qui n'est pas dans nos usages et pourrait nous conduire alors que une procédure. Rapide, avait été adopté à retarder de manière. Totalement inutile l'adoption du texte, je crois que mais, chers collègues, il vaudrait mieux ne pas rigidifier la procédure alors que nous avons déjà suffisamment de garanties sur le délai, dépôt des amendements et sur la date de la séance. Merci, monsieur le rapporteur monsieur Leconte pour l'explication de vote. vote. Monsieur présente ce président de la commission des lois, je pense que le le mieux est l'ennemi du bien en la matière, je crois que vous nous feriez courir un risque constitutionnel si nous ne n'adoption pas l'un des amendements proposés, je vous rappelle le l'article 10 du. Nouveau règlement du Sénat donnera un président de groupe, en particulier la possibilité au plus tard le vendredi précédent la semaine au cours de laquelle est examinent le texte en séance. La possibilité de déclarer qu'il y a un retour à la procédure normale, donc le vendredi, on peut tout à fait imaginer que la conférence des présidents et précisé que le le délai pour les amendements sur le lundi matin, ça veut dire que ça donne le week-end, alors vous allez nous dire pour la conférence des présidents, c'est pas l'usage de s'redevenir le week-end, mais c'est peut-être pas non plus l'usage d'un probable vendredi soir que le délai des Adam rendement pour le texte qui sera en séance mais complètement, pas simplement sur les plans que vous avez évoqué complètement réouvert sera nous aurons que quelques heures pour ça, il me semble que vous, en en refusant ces ces amendements, nous nous attaquons notre droit effectif aux amendements dans tous les cas, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut flexibiliser les choses et donné dans ces cas-là, la possibilité à la conférence des présidents de refixer un délai qui permettent aux parlementaires, aux sénateurs d'avoir le temps de présenter des amendements, pas simplement sur ce qui aurait pu être fait lors de la séance de lecture finalement de la décision de la commission, mais dans une dans dans l'homme à partir du moment où la procédure normale est réouverte, nous avons l'ensemble du texte qui doit être possiblement amendé, est ce que vous proposez ne le permet pas dans tous les cas. Merci, cher collègue. Je n'ai au foie, c'est 3 amendements d'abord le 3 avec un avis défavorable de la commission qui est pour.

Nous passons à l'amendement 12 rectifier défendue par monsieur S'il convient d'accélérer la procédure législative en les clauses accord cette réforme ne doit pas aboutir apporter une entrave excessive au droit d'amendement pardon, prévue par la Constitution et qui constitue la principale expression du droit d'initiative du Parlement, y a des examen des projets, des propositions de loi étendant d'ores et déjà très court, il est indispensable de permettre aux parlementaires de réfléchir sur les sujets traités afin de faire avancer le débat sur les points nouveau qui peuvent se présenter en cours de discussion entre l'examen en commission et la séance à la réflexion se poursuit et souvent elle mûrit, et c'est pourquoi le présent amendement élargit le droit d'amendement qui permet, pour permettre l'examen des amendements qui n'ont pas fait l'objet d'un examen en commission, voilà le sens de cet amendement que je vous propose d'adopter le président aura sans doute un bon geste, presque en fin de séance pour adopter pour nous proposer un avis favorable. Merci, cher collègue, avec des arguments comme ça, je ne sais pas si président ne va pas finir par céder. par céder. Sûr que n'abusez pas de ma réputation de tendresse, vous me compliquer la tâche, je ne peux pas émettre un avis favorable à votre amendement et croyez bien que ça me cause un profond chagrin mais votre amendement viderait de toute substance la procédure de la législation en commission en permettant que soit débattu dans l'hémicycle, tous les abonnements qui auraient été rejetée à l'occasion de la réunion de la commission, comment voulez-vous que je puisse le soutenir. Je le regrette l'avis défavorable. Merci Monsieur le le rapporteur vous le merci, cher collègue. L'amendement numéro 30 et défendu par Madame Assassi. Merci Merci monsieur le président, nous estimons que les dispositions du 2ème alinéa de cet article unique limite le droit d'amendement sur les articles examiné en séance publique dans le cas d'une législation commission partielle, en effet, a indiqué, je cite : il ne peut être reçue en sciences aucun amendement remettant en cause les dispositions faisant l'objet de cette procédure,

il apparaît plus conforme à l'esprit, qui semble être celui de la proposition de résolution de ne pas accepter les amendements portant sur les articles aborder en commission et donc c'est l'objet de notre amendement. Si chers collègues, quel est l'avis de la commission. Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, je ne mets donc on voit qu'il est pour l'amendement 30. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adoptée, nous passons à l'amendement 26 qui est également défendue par Madame la Présidente. donc là il surgit, nous estimons que l'examen de la recevabilité d'un amendement portant sur des articles examiné en séance publique, relève de la compétence du service de la séance, c'est ce service qui, selon nous, est le garant d'une cohérence en matière de recevabilité des amendements, car le risque serait d'évoluer vers des jurisprudences à géométrie variable selon les commissions concernées. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. Avec beaucoup d'égard pour les, pour les services de la séance, je dois vous dire que la règle en matière d'appréciation de la recevabilité des amendements, c'est que l'appréciation est faite. Instance politique et non pas par une instance administrative, oui mais vous voulez justement transmettra une instance administrative le soin de s'opposer à ce que des amendements soient débattues en raison de l'recevabilité, moi je préfère qu'on garde notre règle traditionnelle. Qui permet que la. Commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des amendements, c'est mieux pour nous de conserver cette responsabilité politique, l'avis est défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, je n'aime ou on voit l'amendement avec un avis défavorable de la commission qui est pour,

Quel est l'avis de la commission. examinons ce texte avec la procédure de législation, ça serait pas cohérent, il faut savoir ce que vous voulez donc avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, je mets au voilà maintenant avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas nous arrivons à 3 amendements identiques d'abord le 28 rectifier défendue par monsieur. Merci monsieur le président, mes chers collègues, nous avons, nous, avouant avoir découvert avec autant de preuves que la présente proposition de résolution accompagné la sacralisation du débat en commission par une réduction du temps de parole pour les explications de vote en séance publique, en effet, l'expérimentation qui viennent de se terminer, le train de septembre dernier, dénommé procédure d'examen en commission Estoril, explications de vote de 7 minutes pour les groupes, curieusement, vous nous proposez de réduire ce temps alors que vous appelez de votre voeu une extension de cette nouvelle procédure de plus douze ouvraient le droit à la conférence des présidents de réduire encore ce temps de parole qui deviendra législation en cas d'explications sur des articles examiné en commission dans le cadre de la législation partielle cette obsession de la réduction du droit d'expression des parlementaires et à notre sol c'est inquiétante d'autant plus qu'une dangereuse course à l'échalote s'est engagé entre le Sénat et l'Assemblée nationale en la matière en quoi réduire quasiment à néant le temps de parole des parlementaires qui ne peuvent étayer le moindre argument politique renforce l'-t-il la démocratie ce genre de disposition n'est pas anodine, elle participe, je le répète au grand travail d'affaiblissement des pouvoirs du Parlement au profit d'un exécutif jugé seul efficace pour agir dans un d'espace mondialisé, je vous remercie.

sa main demande la ce sera ma dernière à tentative décide attendrir le président de la commission des lois, et obtenir sa clémence peut-être l'article unique prévoit que lorsque la procédure de législation commission s'applique sur l'ensemble du texte, le gouvernement et les représentants des commissions d'intervention hier et maximale de 7 minutes lorsque cette procédure ne s'applique le que sur certains articles du texte, leur temps de parole est limité à 5 minutes chacun, c'est de parole se présente demeure insuffisante compte tenu de la technicité de certains sujets et il convient dès lors de leur accorder la possibilité de s'exprimer plus longuement, notamment en raison de cette technicité le présent amendement rétablit, temps de parole telles qu'il était prévu dans la version expérimenté de la procédure, les portant respectivement à 10 et 7 minutes, voilà le sens de cet amendement, qui je suis sûr, va connaître un grand succès.

Il est défendu merci ce président prie de l'excuser ce rapporteur cette fois-ci c'est la bonne défavorable merci n'ai donc on voit l'amendement 28 rectifier avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté même vote pour le 17 même vote pour le 29 également, merci, je mets donc on voit l'article unique. De ce texte qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Nous passons à un amendement 18 sur l'intitulé de la proposition de loi

qui est presque contraire à celui de légiférer plus rapidement, chacun sait l'influence qu'ont acquis certains groupes d'intérêts sur le processus législatif, y compris au stade de son élaboration dans les arcanes ministérielles, une meilleure association de l'autre partie de la société civile des citoyens pourrait également être envisagée plus sérieusement par le biais d'outils numériques que nous avons évoqué les qui sont d'ailleurs déjà en application, y compris dans nos murs, vous l'aurez compris ces remarques visant à montrer que la modernisation de notre procédure législative doit également nous amener à envisager ces perspectives plutôt qu'à se limiter à la question de la rationalisation et de la limitation des temps des débats téléobjectif de l'amendement j'espère évidemment bénéficié la tendresse légendaire du président de la commission des lois. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, le président de la commission des lois défavorables merci Monsieur je mets au revoir l'amendement 18 rectifier venant de faire l'objet d'un avis défavorable de la commission des lois, qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, je vais mettre aux voix à l'ensemble de la proposition de résolution, il y a-t-il des demandes d'explications de vote, monsieur, monsieur Oui merci monsieur le président, Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, monsieur le président de la commission des lois à la suite, enfin de de ce débat, vous avez noté que nous avons soutenu cette proposition de résolution du président du Sénat, mais que les 2 amendements que nous vous avons présenté pour améliorer le texte, n'ont pas eu votre soutien, monsieur le président de la commission des lois, nous avons l'impression que c'est un peu asymétrique mais nous voterons quand même ce texte mais en même temps je vous appelle, j'appelle l'ensemble de nos collègues à bénéficier, à profiter de cette nouvelle possibilité pour renforcer l'initiative parlementaire, et j'espère que dès le début de l'année prochaine les PPL que les groupes déposeront dans leur niche pourront après un accord entre les présidents de groupe, lorsque ce sont des des propositions qui ont vocation vraiment à faire progresser les choses qui sont pas Cleveland sur le plan politique, à ce qu'elle puisse prospérer, de cette manière-là, je crois que de cette manière, nous aurons, nous pourrons démontrer que cette résolution que nous vous allons voter peu permettent de renforcer la capacité parlementaire d'initiative législative et de réellement faire progresser d'à capacité du Parlement, de proposer des lois et de les adopter voilà donc je vous invite maintenant à à utiliser cette nouvelle proposition et j'espère, monsieur le président de la commission des lois que ce soutien sera réelle parce que devant une impression de vous souvenir plus que vous souteniez des propositions d'amélioration du texte. Merci, cher collègue Monsieur Président retailles. Oui, Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier le rapporteur, président de la Commission pour le le travail comme à l'accoutumée, excellente à l'à titre personnel, mais aussi pour ses commissions, je voudrais simplement dire que, avec ce texte, et cette résolution on trouve je pense un bon point d'équilibre et le Sénat, une fois de plus, montre qu'il sait se rénover, il s'est modernisé la procédure législative, nous allons, de toute façon, dans quelques mois et revenir avec la révision constitutionnelle un un Champ sans doute encore plus large, simplement cette résolution montre que nous pouvons nous moderniser dans notre pratique de fabrique de la loi et je voudrais simplement dire aux collègues qui sont un peu plus réticents que ce qui est prévu avec non pas un, mais même 2 double droit de véto aux 2, moment crucial où notamment à la conférence des présidents, ce devra être autorisé, ex-santé et puis ensuite, après le travail de la commission Expo, je pense que ce double droit de véto offrent toutes les garanties nécessaires pour que cette nouvelle pratique ne tolère aucune dérive, donc je pense que notre groupe dans son ensemble, et même au-delà de ce que j'ai cru longtemps, nous voterons cette résolution. Merci, cher collègue, monsieur sueur pour explication de vote. Monsieur le le président partageons complètement les propos de Jean-Yves Leconte je voulais ajouter quelques mots monsieur le président, pour le réjouir, comme l'a fait monsieur Retailleau du fait qu'il est là, année les moments de modernité qui nous permet de prendre en compte une évolution qui existe dans de nombreux autres parlements qui donne plus de place aux commissions dans le travail législatif et dans le processus d'adoption des lois, les garanties nécessaires existent puisque, en effet, il suffit qu'un seul groupe soit opposés à la procédure pour qu'elle ne puisse pas être mis en oeuvre, mais je voulais intervenir pour dire que cela ne doit pas, à mon sens, sa secrétaire, dans une logique que je vois prospérer dans un certain nombres de déclaration selon laquelle il faudrait aller plus vite, toujours plus vite et simplifier la procédure toujours davantage ainsi cette idée qu'il serait souhaitable que la procédure accélérée de vin, la procédure de droit commun, je dois vous dire, Monsieur le Président, que je suis totalement opposé à cette idée parce que le temps de la loi mérite toute l'attention tout le travail tout le temps tamis des différentes lectures afin que la loi que nul ne peut être ignoré soit peaufiner préciser notamment ligne après ligne, afin que nous fassions notre travail de législateur l'idée que la précipitation serait une bonne chose est une négation du travail du législateur et le temps de la loi n'est pas forcément le temps de l'exécutif, mais c'est le temps qu'il faut pour que la démocratie fonctionne en donnant au Parlement tout le rôle qui est le sien dans l'intérêt public et dans l'intérêt de la nation, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, cher collègue Madame Assassi

au nom de mon groupe, j'ai défendu un certaine nombre d'amendements qui ont eu des succès d'estime, à défaut d'avoir été adopté mais je pense qu'ils ont nourri alimenter le débat, il enrichit peut-être sans doute est permis peut-être président de d'affirmer de préciser, donner un certain nombre de précisions sur ce texte, somme toute, quand même complexe me féliciter et le j'avais tué le suspense puisque la la discussion générale, j'avais annoncé qu'on groupe votre le texte dont nous le voterons bien sûr même s'il n'a pas été amendé, comme nous le souhaitions, nous serons bien sûr vigilants sur son application, je crois qu'il est un signe de modernité, je m'associe d'ailleurs aux aux propos de Jean-Pierre Sueur sur sur ce point, nous voterons tout simplement ce texte, l'ensemble du groupe RDSE merci. Merci, cher collègue, je mets, on voit l'ensemble de la proposition de résolution, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur l'ensemble de la proposition de résolution, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos, j'invite les secrétaire à procéder au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin numéro 45 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs du groupe politique et notifié à la présidence Nombre de votants : 339 Nombre de suffrages exprimés 339 pour l'adoption 324 contre 15. Le Sénat a adopté. Je vais suspendre la séance, non sans vous avoir remercié spécialement Madame Tremblay, elle sera la séance a repris va 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, puis à 18 heures 30 pour la discussion générale du projet de loi de finances rectificative pour 2017, la séance est suspendue.